La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

unanime au sein de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Nous pouvons nous féliciter de cet accord, qui

bref, à ce qui est aujourd'hui perçu comme un Far West de la consommation, dans lequel les plus vulnérables sont ciblés et l'impunité semble demeurer la règle. Dans un contexte de fortes dénonciations des pratiques d'influenceurs peu scrupuleux, et face à l'agitation médiatique suscitée par les déclarations de diverses personnalités publiques, le Sénat a tenu à travailler en toute indépendance, en entendant toutes les parties prenantes, sans stigmatisation ni préjugés. avions deux objectifs : mieux comprendre le secteur de l'influence commerciale, afin de déterminer le niveau de régulation adéquat pour une activité commerciale en plein développement, et offrir aux internautes et consommateurs, notamment aux plus jeunes d'entre eux, un niveau de protection suffisant.

quels que soient les bénéfices et contreparties qu'ils reçoivent en échange de leurs publications, tout en distinguant leur activité des autres formes de publicité plus traditionnelles. Ces influenceurs seront désormais obligés d'afficher le caractère publicitaire ou commercial d'une publication, en indiquant clairement les mentions « publicité » ou « collaboration commerciale », afin d'éviter la publicité dissimulée et de lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales trompeuses.

régulatrices. L'action des pouvoirs publics devra ainsi être consolidée par le renforcement des pouvoirs de police administrative de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par l'accroissement des moyens d'action de l'Autorité des marchés financiers (AMF), concernant, en particulier, les promotions d'offres illicites sur les réseaux sociaux. Dans ce Far West de la consommation,

niveaux. Il était indispensable de ne pas pénaliser, par exemple, les acteurs du commerce en ligne ou la filière française des crypto-actifs. Les corrections apportées par le Sénat sur ces sujets ont toutes été conservées. ce texte permet, de manière inédite et significative, de renforcer la protection des consommateurs, des internautes, des épargnants, de nos jeunes

l'interdiction de la promotion des conseils ou prestations de pronostics sportifs, l'obligation d'afficher une mention d'interdiction aux personnes de moins de 18 ans pour promouvoir des jeux d'argent

merci de l'engagement des parlementaires et bravo pour la qualité de ce travail ! Il y a quelques mois, des parlementaires de différents groupes politiques exprimaient leur souhait de travailler ensemble sur l'encadrement de l'influence commerciale.

Ce travail conjoint a permis de donner naissance à une proposition de loi précise, ambitieuse et sans précédent en Europe. Sans entrer dans le détail

au sein du processus d'élaboration par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) du référentiel que devront respecter les mécanismes mis en place par les plateformes, afin de soustraire les publics mineurs aux publicités relatives aux jeux d'argent et de hasard. Comme vous le savez,

la commission mixte paritaire conclusive concernant la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux nous permet enfin de fixer précisément le cadre dans lequel la profession encore naissante d'influenceur va devoir évoluer.

Cela étant, en légiférant de cette manière, nous ne stigmatisons pas les influenceurs. Au contraire, nous permettons la restauration de la confiance dans ce secteur, qui a connu des déboires importants ces derniers mois.

par la DGCCRF. Nous mettons aujourd'hui en place un cadre précisant les droits et les devoirs des 150 000 influenceurs français tout en protégeant les consommateurs. Rappelons que, chaque année, plus de 40 millions de nos compatriotes effectuent au moins un achat en ligne.

notion de « mise en relation », nous évitons les effets délétères d'une définition trop large. Nous reconnaissons ainsi leur rôle, alors que la structuration du secteur semble actuellement passer par une organisation cavalière des agents et des agences d'accompagnement des influenceurs. Ensuite, la précision des règles applicables, notamment les rappels formulés à l'article 2 A, ainsi que les interdictions spécifiques à l'influence commerciale, définies à l'article 2 B, viennent répondre aux imprécisions et aux angles morts

Enfin, avec ce texte, nous renforçons l'information du consommateur : la réglementation à venir protégera la jeunesse des publicités agressives pour les jeux d'argent, tandis que l'obligation d'apposer des mentions telles que « publicité » ou « collaboration commerciale » permettra de mettre les points sur les i.

à vous remercier

Face à l'influence croissante des créateurs de contenus, en particulier auprès des jeunes, nous avons souhaité répondre aux préoccupations légitimes suscitées par certaines dérives, telles que la promotion de produits dangereux ou trompeurs, ou simplement de produits ne respectant pas certaines règles éthiques. objectif est de faire passer le message suivant : sur les réseaux sociaux, tout n'est pas permis ! Si nous pouvons regretter que la droite sénatoriale et le Gouvernement aient abordé ce texte sous l'angle

pour davantage de transparence ; l'inscription dans la loi d'un cadre très strict régulant la promotion des produits de santé ; enfin, le rappel de l'obligation d'afficher les normes qui s'appliquent aux boissons et aux produits alimentaires trop gras, trop salés, trop sucrés- une mesure à laquelle notre collègue socialiste, Dominique Potier, a contribué et que nous étions nombreux à défendre sur ces travées. À l'heure de conclure nos débats, rappelons que l'aboutissement de ce texte doit

les sujets du harcèlement et des arnaques en ligne, ainsi que, plus généralement, de la sécurisation de l'espace numérique. En attendant, nous pouvons nous féliciter collectivement de créer le premier cadre en Europe pour réguler l'influence commerciale.

citoyen et écologiste. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre économie connaît de nombreuses évolutions, intensifiées par l'essor du numérique et des réseaux sociaux. De nouvelles formes d'activités émergent, et avec elles de nouvelles habitudes de consommation et de publicité. Nos logiciels de régulation et de contrôle des pratiques commerciales, pensés pour les activités physiques, doivent évoluer et s'adapter à ces nouvelles configurations, sous peine de devenir obsolètes. L'activité d'influence sur les réseaux sociaux s'est développée à une vitesse fulgurante, prenant de multiples formes et touchant de nombreux domaines : mode de vie, cuisine, mode, jeux vidéo, sport ou encore musique. Tous ces secteurs ont vu émerger des créateurs de contenus, qui sont devenus de véritables supports publicitaires pour les marques qui les sollicitent. L'intérêt commercial est évident est évident : ces influenceurs fidélisent des communautés d'abonnés qui les suivent au quotidien, qui les considèrent parfois comme des modèles et qui, de fait, se fient à leurs propos, tiennent compte de leurs conseils et adoptent leurs comportements. Cette confiance est un excellent levier pour transformer l'abonné en consommateur, plus efficace encore que la bonne vieille publicité entre deux dessins animés ou au milieu d'un film. C'est désormais dans les contenus de votre influenceur préféré que le produit vous est vanté que réside tout l'enjeu de la régulation de ce secteur : un besoin de clarté, de lisibilité et d'information, toutes qualités qui sont loin d'être la norme dans le milieu de l'influence sur les réseaux sociaux. Certains de ses acteurs font preuve d'exemplarité et mentionnent systématiquement leurs partenariats rémunérés ; d'autres, au contraire, omettent de le préciser et font passer cet acte commercial pour un conseil de bonne foi sans intention particulière.

: l'introduction d'une responsabilité solidaire entre les influenceurs et leurs agents en cas de dommages causés aux tiers ou encore la soumission de leur relation à un contrat de droit français, dès lors que le public ciblé réside sur le territoire français.

De même, l'instauration d'une représentation légale sur le territoire européen apparaît comme un moyen efficace de mettre un terme à l'impunité qui, jusqu'ici, permettait à certains de multiplier les abus et les pratiques déloyales. Cela dit, nous souhaitons rappeler l'importance de doter ce texte des moyens nécessaires à son application. Les effectifs de la DGCCRF seront au coeur du contrôle de la régulation des activités d'influence. Or, en l'état, cette proposition de loi risque de ne pas pouvoir se concrétiser. Nous l'avons dit durant les débats et nous le répétons ici

Il est temps désormais de réfléchir à la publicité dans son ensemble et d'interdire enfin la promotion de ces produits alimentaires sur l'ensemble des supports. Nous sommes prêts à travailler sur cette

mes chers collègues, alors que les innovations numériques des dernières années ont complètement bouleversé le monde du travail, toutes les composantes de l'ère 2.0 ne sont pas forcément bonnes à prendre. Sur les réseaux sociaux, des dérives parfois dangereuses pour les internautes font surface L'expansion de l'espace numérique permet en outre l'apparition de personnalités dites publiques qui méconnaissent ou ne respectent pas les règles commerciales.

Les influenceurs promeuvent tout, et bien trop souvent n'importe quoi, auprès de leur public. Les jeunes sont plus perméables aux influences, et ils ne sont pas toujours en mesure d'évaluer les risques que celles-ci leur font courir. Ces promotions, parfois anodines et attractives, peuvent très vite devenir dangereuses pour la santé où se révéler être de véritables escroqueries. Comme cela a été rappelé durant les débats en première lecture, des pratiques néfastes pour la santé sont promues sans le moindre encadrement. Elles concernent, entre autres, les produits de beauté, la chirurgie esthétique ou encore des pratiques visant à perdre du poids, tout cela sans l'avis d'un professionnel de santé. Le champ des dangers est vaste. On peut y ajouter les incitations à jouer à des jeux vidéo, à des jeux d'argent ou les conseils relatifs à l'entrepreneuriat et à la finance. Certains influenceurs se retrouvent ainsi vecteurs de l'addiction ou de l'escroquerie. Derrière ces dérives, une rémunération, souvent excessive, atteignant parfois des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, fait oublier à l'influenceur, consciemment ou non, les conséquences de ses actes. phénomène, les mesures législatives actuelles sont bien trop limitées et inadaptées pour prévenir et sanctionner les abus. Une régulation s'impose donc rapidement afin de préciser la responsabilité de l'influenceur dans sa pratique commerciale et de protéger les internautes. De fait, De fait, le RDSE salue l'initiative des auteurs de la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur tous les réseaux sociaux, au même titre qu'il se réjouit que la CMP fût conclusive.

Souhaitons que cela couvre totalement les contenus proposés par ces influenceurs. La rédaction de compromis de l'article 1, qui définit l'activité d'influenceur, inclura bien les avantages accordés en nature ; c'était l'un des souhaits de mon collègue Henri Cabanel. Le renforcement de l'encadrement des publicités autour de la santé publique, notamment l'intégration des dispositifs médicaux de diagnostic, est également une bonne chose. Enfin, attentifs à la lutte contre les addictions, nous sommes favorables au compromis trouvé par nos deux assemblées concernant l'interdiction, pour les personnes exerçant une activité d'influence commerciale par voie électronique, de faire la promotion d'abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, ainsi que des jeux d'argent ou de hasard. Mon collègue Henri Cabanel l'a rappelé en première lecture, l'influence est devenue un métier sans état d'âme. Compte tenu de la réalité alarmante des dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, le RDSE confirme son souhait de voir aboutir ce texte, qui encadrera la profession afin de mieux protéger nos concitoyens, en particulier les plus jeunes et les plus fragiles. La parole est Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chère Amel, mes chers collègues,

car si le droit s'arrête parfois aux frontières, les activités numériques s'affranchissent de celles-ci et les traversent avec aisance et rapidité, de manière parfois déconcertante pour les législateurs que nous sommes. que nous sommes. Nous devons donc tous oeuvrer pour un meilleur encadrement de nos usages et de nos pratiques numériques. Lors de l'examen du texte en commission, nous avons adopté une logique claire, dont je me félicite qu'elle ait été conservée,

Ces créateurs de contenus sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Au niveau mondial, le marché de l'influence est estimé à plus de 32 milliards de dollars. C'est vertigineux Le Parlement a souhaité réguler cet emploi naissant, sujet à toutes les dérives. Instagram est le réseau social de référence, mais d'autres réseaux en accueillent chaque jour davantage, à l'image de TikTok. Ces influenceurs nouent parfois des partenariats avec des marques, et ils publient alors des contenus promotionnels. Si l'immense majorité des influenceurs respectent la loi et ont connaissance du cadre réglementaire, en échange de contreparties en nature ou financières, peuvent abuser de la confiance de ceux qui les suivent, en particulier les plus jeunes. Ces créateurs de contenus malhonnêtes, qui sont parfois appelés « influ-voleurs », pénalisent l'ensemble de la profession. Cette proposition de loi s'attelle à ce vaste chantier et apporte un encadrement bienvenu. Le texte a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 mars 2023, puis par le Sénat le 3 mai dernier. Il s'agit d'une proposition de loi transpartisane, un indicateur positif dont nous pouvons nous réjouir. Il témoigne du vaste consensus qui entoure la régulation de ces activités naissantes. Je me réjouis que la commission mixte paritaire soit parvenue à une rédaction commune sur l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi la définition du métier d'influenceur retenue dans le texte allie une partie de la rédaction proposée par le Sénat et une partie de la rédaction issue de l'Assemblée nationale. Ce compromis montre bien l'esprit de collaboration qui a animé les échanges depuis le début. C'est une bonne chose.

afin de protéger les consommateurs, les mineurs. Nous devons conforter et « muscler » le cadre réglementaire. La proposition de loi rappelle le cadre juridique existant. Elle permet de l'expliquer avec pédagogie et de le contrôler pour éviter les dérives. Les modifications issues des échanges en commission mixte paritaire vont dans le bon sens. Nous l'avons rappelé, ce travail est inédit au sein de l'Union européenne. Par ce texte unique en son genre, nous ouvrons une voie nouvelle. Nous pouvons être fiers de cette première pierre apportée au défi de la régulation

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous saluons le travail accompli ces derniers mois par les auteurs du texte et les rapporteurs des deux chambres. Nous votons aujourd'hui un texte attendu, qui vise à réguler l'influence commerciale et à responsabiliser un secteur en voie de structuration. Le marché mondial du marketing d'influence a atteint 15,5 milliards d'euros en 2022, soit +20 % en un an. Instaurer un cadre réglementaire et fixer un certain nombre de règles pour réguler cette activité en pleine expansion était donc nécessaire. Si une grande part des acteurs exercent leur activité avec honnêteté, certains ignorent, voire s'affranchissent des règles de base du commerce et de la publicité. Des abus, et parfois des escroqueries ont bien lieu.

sens. Nous regrettons toutefois fortement que la promotion d'un certain nombre de produits ou de pratiques, qui nous paraissent particulièrement nocifs pour la santé physique et mentale de la jeunesse, ne soit pas interdite ou, tout du moins, drastiquement encadrée.

Nous restons convaincus par les alertes des scientifiques et des organismes de santé comme l'OMS ou Santé publique France. Au regard des risques cardiovasculaires, de surpoids et de diabète qu'induit une alimentation basée sur des produits de faible qualité

produits. Mon groupe est consterné par le maintien de la suppression de l'article 2 CA, qui visait à interdire aux enfants de moins de 16 ans exerçant l'activité d'influence commerciale de faire la promotion de ces produits alimentaires et des boissons trop riches en sucre.

Celle-ci envahit nos imaginaires, incite à surconsommer, des produits polluants. La réclame a sa part de responsabilité dans la crise écologique et dans cette forme de malaise et de frustration qui peut imprégner notre jeunesse. Elle devrait être enfin mieux encadrée.

Il nous paraît primordial d'interdire l'exposition de nos adolescents à la promotion de traitements, hors contexte médical, qui ne leur conviennent pas nécessairement et peuvent avoir des conséquences graves, parfois irréversibles, sur leur apparence physique et leur santé. Malgré ces points problématiques, le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires votera ce texte. Si ce dernier manque un peu d'ambition, il a le mérite de poser une première pierre pour que cet écosystème assez hétérogène agisse de manière responsable, éthique et respectueuse de son public. Je souhaite également saluer votre engagement,

Le scrutin est clos.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Par ailleurs, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.

visant à interdire l'importation de produits issus du travail forcé de la population ouïghoure en République populaire de Chine, présentée par Mme Mélanie Vogel, M. Guillaume Gontard et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 242).

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur l'initiative de notre collègue Mélanie Vogel, qui regrette de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui et qui vous prie de bien vouloir l'en excuser, le groupe Écologiste-Solidarité et Territoires propose que le Sénat s'exprime à son tour sur l'indicible crime contre l'humanité opéré méthodiquement depuis plus de dix ans dans l'ouest de la Chine. Pour compléter la résolution portant sur la reconnaissance nous vous proposons, de manière plus opérationnelle, de stopper l'importation des produits issus du travail forcé des Ouïghours, en France comme en Europe. en Europe. Grâce à la mobilisation de tous les instants de la diaspora ouïghoure, relayée notamment par notre collègue député européen Raphaël Glucksmann, nous savons beaucoup du traitement inhumain dont est victime la minorité ouïghoure de Chine. Chine. Permettez-moi néanmoins de rappeler une nouvelle fois l'ampleur de l'horreur qui est à l'oeuvre dans le Xinjiang. Depuis le début des années 2010, et surtout depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping, la République populaire de Chine mène une stratégie d'assimilation culturelle violente envers les groupes minoritaires, particulièrement envers la minorité musulmane ouïghoure dans la région autonome du Xinjiang. Cette politique d'épuration ethnique se traduit par l'interdiction de pratiques religieuses et culturelles, la destruction de lieux de culte et de cimetières religieux ou encore la surveillance de masse. Les autorités chinoises font tout ce qui est en leur pouvoir pour diminuer la présence de l'islam, transformant le Xinjiang en laboratoire de la politique d'assimilation répressive du parti communiste chinois. Sous couvert de lutte antiterroriste, le gouvernement chinois criminalise toute expression des traditions. Sous couvert de lutte contre l'extrémisme religieux, le gouvernement chinois s'octroie le droit d'incarcérer dans des camps de rééducation toute personne qui pratique la religion musulmane. La pratique du ramadan, la consommation de nourriture halal, une apparence jugée trop religieuse ou encore l'enseignement coranique suffisent à vous envoyer dans un camp de rééducation, où les détenus sont forcés d'abandonner leur religion. Et pour le prouver, les autorités chinoises forcent les détenus à boire de l'alcool, à manger du porc ou encore à prêter allégeance au parti communiste chinois. D'autres témoignages issus de ces camps, notamment de femmes kazakhes ou ouïghoures, font froid dans le dos. Il y est fait état d'abominables contrôles des naissances se traduisant par la pose contrainte de contraceptifs, des avortements et des stérilisations forcées.

Au milieu des années 2010, les arrestations préventives et les placements dans des camps se multiplient, sous des prétextes de plus en plus dérisoires, comme une simple discussion avec un résident étranger. Les incarcérations se font, naturellement, en dehors du système judiciaire. Des dispositifs de surveillance massive sont mis en place pour traquer les musulmans. Des fonctionnaires sont envoyés vivre dans les familles musulmanes pour surveiller leur mode de vie, ce qu'elles mangent ou la manière dont elles éduquent leurs enfants. Une vaste politique de délation, qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité, est promue par les autorités chinoises. Les Ouïghours sont également traqués à l'étranger, les autorités chinoises leur demandant des informations sur le reste de la diaspora et les menaçant de s'en prendre à leur famille restée en Chine s'ils refusent de répondre. C'est en 2017 que les premières preuves de l'existence de ces camps émergent et que les premières réactions internationales se font entendre. Amnesty International et l'Organisation des Nations unies estiment qu'il existe 1 200 camps de rééducation au Xinjiang, et que 1 million de prisonniers y sont incarcérés, Quelques mois plus tard, l'on découvre que le gouvernement chinois organise un système de travail forcé des Ouïghours. Dans un rapport des autorités chinoises datant de 2020, nous apprenons que 2,6 millions de citoyens ouïghours du Xinjiang ont été placés dans des fermes et des usines. Un système organisé au plus haut niveau permet aux industriels de passer des commandes de travailleurs aux autorités locales. Des recruteurs sont désignés et des quotas de travailleurs à atteindre, fixés. Ils se rendent au sein des foyers pour recruter des travailleurs. Tous les habitants turciques de plus de 16 ans sont susceptibles d'être forcés d'aller travailler et sont menacés de détention. Pendant quelques jours, ils sont formés à des tâches répétitives, puis ils sont envoyés dans les usines. Ils sont entassés dans des dortoirs, ne peuvent pas démissionner, travaillent pendant un nombre incalculable d'heures en contrepartie de très bas salaires.

encore les panneaux solaires. Disons-le clairement : c'est toute une partie de l'appareil industriel chinois auquel nous avons délégué la production de tant d'objets de notre quotidien qui repose sur le travail forcé, comme en son temps, la production industrielle soviétique. Notre attitude était alors tout autre.

le 31 août 2022, dans un rapport accablant, résultat de sa visite dans le Xinjiang. Les conclusions de ce rapport sont sans appel : elles confirment toutes les révélations des associations de défense des droits de l'homme. Malgré les nombreuses réactions internationales, très peu des marques mises en cause ont répondu aux accusations, et celles qui ont arrêté de faire appel aux usines du Xinjiang se comptent sur les doigts d'une main. mes chers collègues, les indignations ne suffisent plus. Leur coût politique et économique est bien trop faible. En 2021, le commerce direct entre le Xinjiang et l'Union européenne a même augmenté de 13,6 %. C'est tout un système économique mondial fondé sur le profit et l'exploitation de la vie humaine qu'il faut combattre. Aujourd'hui, on sait qu'un vêtement sur cinq porté sur la planète peut être entaché de travail forcé ouïghour. C'est vertigineux L'Europe doit prendre ses responsabilités. Nous avons le devoir de nous doter d'une politique commerciale exigeante respectant les droits humains les plus basiques. Les initiatives dans ce sens se multiplient, et la France, qui se veut le phare de la promotion des droits partout dans le monde, doit produire son effort et son effet. En 2021, les États-Unis ont interdit d'importer des produits fabriqués dans la province chinoise du Xinjiang. Tout produit fabriqué, même partiellement, dans le Xinjiang, est considéré comme étant issu du travail forcé et ne peut être importé, sauf si les entreprises sont en mesure de fournir des preuves claires et convaincantes du contraire. Dans le même esprit, la Commission européenne a présenté au mois de septembre dernier un projet qui permettrait, à terme, d'interdire certains produits d'entrée sur le marché européen. En cas de soupçons sur un produit, les organismes chargés de la surveillance des marchés pourront lancer une enquête préliminaire au terme de laquelle le produit soupçonné pourra être banni du marché européen. des motifs de cette proposition de résolution, nous souhaiterions que la France et l'Europe adoptent une position proche de celle des États-Unis. Nous pensons en effet que la charge de la preuve doit être inversée ce sont les industriels qui doivent prouver de manière convaincante qu'ils ne se fournissent pas dans des usines faisant appel au travail forcé des Ouïghours. Ce ne sont pas aux pouvoirs publics ou aux lanceurs d'alerte d'en apporter les preuves. Je précise au passage qu'adopter la position américaine en la matière n'est pas du tout synonyme, dans notre esprit, d'un alignement complet avec les positions américaines dans la guerre commerciale, parfois quelque peu manichéenne, engagée contre la Chine. Au regard des bouleversements géopolitiques majeurs que nous connaissons ces dernières années, l'Europe et la France sont dans la nécessité impérieuse de redéfinir leurs relations avec la Chine et de construire une politique chinoise qui nous soit propre. tenu des valeurs portées par notre pays et notre union continentale, la fermeté absolue vis-à-vis des crimes contre l'humanité doit à nos yeux constituer une composante essentielle de notre relation avec Pékin. Alors que l'Assemblée nationale a adopté au mois de janvier 2022 une proposition de résolution portant sur la reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques systématiques, ainsi que des crimes contre l'humanité actuellement perpétrés par la République populaire de Chine à l'égard des Ouïghours, comment pouvons-nous continuer à importer, vendre et consommer des produits qui sont fabriqués dans des conditions de travail forcé n'ayant pas grand-chose à envier au goulag ? il est plus que logique et cohérent de demander au Gouvernement d'adopter des mesures efficaces pour cesser, selon les mots de notre collègue Mélanie Vogel, « d'offrir un débouché commercial aux crimes contre l'humanité En mettant en place une politique qui rejette tout produit issu du travail forcé des Ouïghours, la France ferait peser une vraie chape de plomb sur la Chine, qui mise énormément sur le développement du Xinjiang, région qui est au coeur du projet de nouvelle route de la soie du fait de sa situation géographique, au croisement de routes commerciales entre les continents européen et asiatique. Le seul rapport de force que comprend la Chine est économique, et c'est à son portefeuille qu'il faut s'attaquer pour tenter de retrouver le sens de notre humanité. La

proposition de résolution. Depuis 2017, des millions d'Ouïghours et membres d'autres minorités musulmanes ont disparu dans un vaste réseau de camps de rééducation dans la région du Xinjiang. programme de génocide culturel mené par le gouvernement chinois : des femmes subissant des stérilisations forcées ; des détenus soumis à un endoctrinement politique, contraints de renoncer à leur religion, à leur culture, soumis à la torture.

dans les secteurs de la technologie, de l'industrie et, surtout, de la mode, a mis au jour l'utilisation massive par de grandes marques du système concentrationnaire mis en place au Xinjiang par la République populaire de Chine. Que s'est-il passé depuis ? Quelques marques, comme Adidas ou Nike, ont annoncé avoir cessé de s'approvisionner au Xinjiang ; certaines, comme Zara ou Hugo Boss, ont condamné ce système, avant de revenir sur leurs déclarations pour ne pas froisser en Chine ; beaucoup d'autres sont simplement restées silencieuses. Dans les faits, rien n'a changé. Les associations, comme Sherpa ou l'Institut ouïghour d'Europe, ont déposé de nombreuses plaintes, mais 20 % du coton mondial est toujours produit dans la région autonome du Xinjiang. même de cet hémicycle, aujourd'hui, les vêtements que nous portons, les téléphones dans nos poches, les écrans sont très certainement produits en partie au prix de la liberté d'un peuple réduit en esclavage. Le système de traite des êtres humains mis en place contre les Ouïghours est un moteur de la politique industrielle industrielle de la République populaire de Chine, le carburant sanglant de la stratégie commerciale des nouvelles routes de la soie du gouvernement de Pékin. Un million, ou plus probablement deux millions de personnes sont enfermées dans des camps de travail, enfermées et torturées, parfois simplement pour avoir parlé leur langue dans la rue ou pour appelé quelqu'un à l'étranger. On parle ici de 10 % de la population ouïghoure. Aujourd'hui, les sénateurs peuvent regarder les yeux grand ouverts la réalité que le régime chinois veut masquer, étouffer, nier : nous sommes face à la plus grande campagne d'internement d'une population depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, que fait concrètement la France ? Trop peu, hélas ! Bien sûr, symboliquement, l'Assemblée nationale a reconnu par une résolution l'année dernière qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité, et nous le saluons. Mais après ? Rien ne fait vraiment obstacle à la circulation en Europe des produits issus du travail forcé. Aujourd'hui, nous vous invitons à avancer sur cette question fondamentale en demandant au Gouvernement français de travailler à l'échelle européenne, le plus grand marché mondial, pour mettre en place un véritable mécanisme de contrôle des produits issus du travail forcé en Chine. Nous souhaitons ici nous inspirer de ce que font déjà les États-Unis et le Canada, entre autres États, en inversant la charge de la preuve. Oui, aux États-Unis, depuis l'an dernier, si un produit a été fabriqué, en tout ou partie, dans le Xinjiang, il est considéré comme issu issu du travail forcé, à charge ensuite aux entreprises de prouver le contraire. Résultat : une baisse remarquée des importations en provenance de Chine aux États-Unis, qui, malheureusement, s'est accompagnée dans le même temps d'une augmentation des importations chinoises Il nous faut donc désormais, nous aussi, demander aux entreprises souhaitant accéder au marché commun européen de prouver que la traçabilité de leurs produits est sans reproche. En ce moment même, à Bruxelles, on s'apprête malheureusement à mettre en place le processus inverse, c'est-à-dire un processus long et compliqué, difficilement lisible, qui impose aux États membres de fournir eux-mêmes la preuve du travail forcé pour interdire les produits incriminés. C'est un processus absurde et inefficace : tout le contraire de ce qu'il faudrait faire ! À l'inverse, cette résolution que nous vous proposons d'adopter aujourd'hui relève du bon sens. La représentation nationale a déjà condamné le « caractère génocidaire » des violences à l'encontre des Ouïghours. Soyons cohérents et logiques en traduisant ces intentions dans les actes. Comment dénoncer un crime contre l'humanité sans interdire sur notre sol les fruits de ce crime ? Il y va de l'honneur de la France d'être le moteur, à l'échelle européenne, d'une initiative claire, nette, qui ferait véritablement obstacle à la circulation des produits de l'esclavage moderne. Ce serait un message puissant envoyé à Pékin, mais qui aurait aussi un caractère universel. Le travail forcé

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, je veux tout d'abord remercier le groupe GEST, à l'origine du texte que nous étudions aujourd'hui. En effet, c'est la première fois- je dis bien la première fois -que notre Haute Assemblée est amenée à débattre de l'abominable tragédie qui frappe la frappe la population ouïghoure. Disons-le tout net : il était temps ! Quand, voilà dix ans, j'ai pris l'initiative d'inviter les représentants du Congrès mondial ouïghour dans nos murs, j'avoue avoir ressenti un grand moment de solitude, car rares étaient à l'époque les parlementaires un tant soit peu informés de cet effroyable drame. Depuis, la coercition massive exercée à l'encontre de cette minorité ethnique n'a cessé de s'intensifier, et il aura fallu l'incroyable persévérance de quelques associations et chercheurs pour parvenir à documenter ce que d'aucuns osent désormais appeler un véritable processus génocidaire. Même si le travail forcé ne constitue qu'une des multiples exactions mises en oeuvre par le régime de Pékin à l'encontre des Ouïghours, cette proposition de résolution est aussi l'occasion de parler de cette forme d'esclavage moderne qui est aujourd'hui en forte résurgence en Chine, mais aussi ailleurs dans le monde. La lutte contre ce fléau remonte à 1930, puisque la convention visant à combattre le travail forcé fut parmi les premières adoptées par l'Organisation internationale du travail (OIT) créée en 1919. S'en est suivie l'adoption d'une seconde convention pour l'abolition du travail forcé en 1957. Sur le papier, nous pourrions nous réjouir que la quasi-totalité quasi-totalité des États de la planète aient aujourd'hui ratifié ces deux conventions. Très récemment, le 12 août 2022, la République populaire de Chine a, à son tour, fini par les ratifier, et leur entrée en application dans ce pays est supposée intervenir d'ici à deux mois et demi.

Loin de régresser, le travail forcé connaît une recrudescence très inquiétante depuis le milieu des années 2010. L'OIT estime à 28 millions le nombre de personnes qui en sont victimes dans le monde en 2021, un chiffre en progression de près de 3 millions par rapport à 2016. Pour des raisons très politiques, l'OIT publie non pas des données par pays, mais seulement des agrégats régionaux. Heureusement, nous en savons davantage grâce à la, qui vient de publier son dernier rapport voilà tout juste une semaine. Son index mondial, qui agrège travail forcé, mariage forcé et traite humaine, fait apparaître que la Chine, avec 5,8 millions de personnes soumises à ces formes scandaleuses d'esclavage moderne, se situe au deuxième rang mondial, derrière l'Inde. En Chine continentale, ce chiffre a même connu une progression de 70 % au cours des cinq dernières années. Au contraire de l'Inde, où le travail forcé est plus diffus sur l'ensemble du territoire, le phénomène en Chine est davantage concentré dans des régions comme le Xinjiang ou le Tibet, et il est, comme en Corée du Nord, le fruit d'une politique délibérée de l'État, et non le fait d'acteurs privés, comme dans la plupart des autres pays. Il serait illusoire de croire que la ratification des deux conventions de l'OIT changera les choses en Chine, et au Xinjiang en particulier. Qui sera autorisé à aller sur le terrain vérifier leur application ? Rappelons-nous, mes chers collègues, la tragicomédie de la mission d'inspection de l'Organisation 2021, au laboratoire de virologie de Wuhan. Rappelons-nous le fiasco du déplacement de Michelle Bachelet au Xinjiang en mai 2022. Il y a dix ans, quand la Chine a officiellement aboli la rééducation par le travail, le seul véritable changement a été la requalification sémantique des « camps de rééducation » en « centres de formation professionnelle En réalité, cette ratification par la Chine des conventions de l'OIT est une tentative de fournir un alibi à la Commission européenne pour rouvrir la ratification de l'accord global sur les investissements Union européenne-Chine. Signé en catimini le 30 décembre 2020, celui-ci a été suspendu après le tollé provoqué par les sanctions imposées par à plusieurs eurodéputés défendant la cause ouïghoure. Pour ne pas perdre la face devant l'opinion publique européenne, la Commission tente actuellement de finaliser un règlement interdisant l'importation de produits issus du travail forcé. Mais, en l'état, elle n'est pas dotée des moyens nécessaires pour en assurer la traçabilité effective. La grande faiblesse du texte de la Commission, c'est de faire peser la charge de la preuve sur le régulateur, un régulateur qui a déjà bien du mal à assurer un suivi systématique des accords commerciaux dont il a la responsabilité. L'intérêt majeur de la résolution ici en discussion est précisément de faire porter la charge de la preuve sur les entreprises responsables de l'introduction de ces produits sur le marché européen. Il ne s'agit en rien d'une mesure d'exception. Elle est conforme au droit européen et s'applique déjà dans plusieurs domaines. Pour en terminer, je rappelle que les produits issus du travail forcé consommés en France représentent un chiffre d'affaires annuel de près de 12 milliards de dollars, dont 8

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est des moments où notre chambre a l'occasion de se grandir en laissant une trace dans l'Histoire. Ce fut le cas récemment, avec l'adoption, le 23 mai dernier, du projet de loi relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites entre 1933 et 1945, ou encore avec l'adoption de la résolution relative à la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens au mois de février.

Je veux aussi rendre hommage aux Ouïghours eux-mêmes qui, au risque de leurs vies et de celles de leurs familles, témoignent et informent le monde de ce crime contre l'humanité que subit leur peuple.

Selon une enquête réalisée par le chercheur allemand Adrian Zenz et révélée en 2020, au moins un demi-million d'habitants du Xinjiang issus des minorités ethniques sont envoyés dans les champs de coton pour y travailler de force. Selon l'Organisation internationale du travail : « Le travail forcé fait référence à des situations dans lesquelles les personnes sont contraintes de travailler par l'utilisation de la violence ou de l'intimidation, ou des moyens plus subtils comme l'accumulation de dettes au Xinjiang, les 11 millions d'Ouïghours, de Kazakhs et autres peuples musulmans sont bel et bien soumis à un contrôle policier totalitaire et à un travail forcé. Depuis 2017, des centaines de milliers d'entre eux ont été envoyés en camps de rééducation.

Fin 2018, après avoir longuement nié, la Chine a reconnu l'existence de ces camps, les présentant comme des lieux « sympathiques » de formation professionnelle. Une véritable honte

consacré à la région autonome ouïghoure du Xinjiang concluait que de « graves violations des droits de l'homme » étaient commises à l'encontre des Ouïghours et d'« autres communautés majoritairement musulmanes Déjà, à l'époque, ce rapport affirmait que « les allégations de pratiques de torture ou de mauvais traitements, notamment de traitements médicaux forcés et de mauvaises conditions de détention, étaient crédibles, tout comme les allégations d'incidents individuels de violences sexuelles et sexistes

en être fière. En juin 2022, le Parlement européen adoptait deux résolutions : l'une sur la situation des droits de l'homme au Xinjiang, y compris les fichiers de la police du Xinjiang, et l'autre sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé. Preuve, s'il en fallait, que ces initiatives démocratiques ne laissent pas de marbre le régime de Pékin, celui-ci avait, en représailles, sanctionné une dizaine de ressortissants européens, dont des parlementaires, comme Raphaël Glucksmann.

qu'elle n'est pas suffisante. Le texte que nous examinons aujourd'hui, lui, va dans le bon sens, puisqu'il invite les instances européennes à réviser cette proposition en s'inspirant des dispositions mises en oeuvre par les États-Unis, qui interdisent les produits et font peser la responsabilité

Il faut le savoir, chacune et chacun d'entre nous, chaque personne qui porte un vêtement ou un accessoire qui comprend, à un moment ou à un autre de sa chaîne de production, une fibre de coton produite en Chine, doit envisager la forte probabilité d'être bénéficiaire, à son insu, du travail forcé d'Ouïghours.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux commencer en remerciant le groupe GEST de la proposition de résolution visant à interdire l'importation de produits issus du travail forcé de la population ouïghoure du Xinjiang. À notre tour, sans réserve et fermement, nous condamnons les crimes de masse commis à l'encontre de cette population. Le rapport issu de l'enquête du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU présente des éléments probants travail forcé, séparation des familles, camps de travail, application brutale et discriminatoire de la politique de contrôle des naissances jusqu'à la stérilisation forcée, torture, viols. Il n'utilise cependant pas encore le qualificatif « génocidaire », contrairement à la résolution que nous examinons aujourd'hui. Vous connaissez nos réserves quant à l'utilisation de ce terme tant que l'ONU n'a pas statué officiellement. Il n'en reste pas moins que ce rapport et les nombreuses enquêtes journalistiques suffisent à conforter notre condamnation de la répression de masse conduite à l'encontre de la population ouïghoure. Nous appelons d'ailleurs la Chine à permettre une enquête indépendante sur son territoire Si ces crimes sont à examiner dans le cadre de l'ONU, les États ne doivent pas pour autant rester silencieux. Cette résolution s'attaque à un volet qui peut être décliné aux échelons national et européen : l'interdiction de produits issus du travail forcé de la population ouïghoure en Chine. Mes chers collègues, dans la fraternité humaine et la solidarité, il ne peut y avoir ni tri ni deux poids, deux mesures. Notre groupe, comme toujours, condamne toutes les oppressions, violences ou crimes commis contre un peuple ou une minorité non seulement les exactions commises à l'encontre des populations ouïghoures, mais aussi celles qui sont infligées aux Palestiniens par la colonisation israélienne, aux Sahraouis, toujours niés par le pouvoir marocain, au peuple cubain, qui subit un blocus américain insupportable, aux Rohingyas, victimes de persécutions en Birmanie.

De plus, la référence à la résolution américaine promulguée par Biden en 2021, dans la foulée des sanctions de Trump, est problématique. Les décisions états-uniennes s'inscrivent dans une logique de guerre économique bien éloignée des droits humains, qu'ils ne se privent pas de fouler en bien d'autres occasions, partout sur la planète, et notamment au Moyen-Orient. La lutte contre le travail forcé ne doit ni connaître de frontières ni devenir l'instrument à géométrie variable des guerres économiques. Le travail forcé n'advient pas uniquement dans les camps du Xinjiang. D'après les chiffres de l'OIT, il concerne plus 27 millions de personnes, hommes, femmes et enfants, sur la planète. Par ailleurs, trop de populations sont exploitées pour des salaires de misère, qui ne suffisent pas à vivre dignement. 50 millions de personnes vivent dans des situations d'esclavage moderne. Aucune région du monde n'est épargnée. L'Asie et le Pacifique comptent plus de la moitié du total mondial, avec 15 millions de travailleurs forcés, l'Europe et l'Asie centrale ne sont pas en reste, avec près de 4 millions, et 3,8 millions de personnes sont concernées en Afrique. Depuis 2017, la situation mondiale se dégrade. La pandémie de covid-19, les conflits armés, le changement climatique, les atteintes graves aux droits humains exposent les populations au risque d'exploitation débridée. Surtout, il ne faut pas oublier que trop de multinationales s'en rendent coupables. Attirées par la logique du profit maximal, elles trouvent leur compte dans les États autoritaires et dans le moins-disant social et environnemental. Dénonçons dès lors toutes les situations de travail forcé, qui font système dans un monde ravagé par l'argent-roi et qui apparaissent avec les traités de libre-échange inspirés par nos logiques commerciales. Dénonçons à raison ce qui se passe non seulement en Chine, mais aussi au Moyen-Orient, singulièrement au Qatar, ainsi que l'enfer des 40 000 enfants travaillant dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Interrogeons nos modes de production et de consommation, socialement et écologiquement irresponsables. Pour lutter efficacement contre le fléau du travail forcé, exigeons des certifications des entreprises sur leurs chaînes d'approvisionnement. Des secteurs sont cités avec insistance dans le rapport de l'OIT : agriculture, mines, industrie manufacturière ou construction. Mes chers collègues, même si nous avons une divergence sur l'évolution restrictive du règlement européen, qui en réduirait la portée potentiellement universelle, le groupe CRCE, à l'exception

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous avez certainement entendu parler de Shein, allégorie de la : t-shirts à 2 euros, robes à 9 euros et accessoires de mode défiant toute concurrence. Tel est le prix de l'esclavage moderne. Le 5 mai, cette enseigne chinoise a ouvert en plein coeur de notre capitale, et pour la seconde fois, une boutique éphémère, où des milliers de Français se sont précipités pour effectuer des achats. À qui pouvons-nous jeter la pierre ? Au consommateur, qui, faisant face à l'inflation, souhaite acheter à moindre coût, ou au Gouvernement, qui permet que ce géant chinois exploitant les Ouïghours comme main-d'oeuvre forcée s'installe librement sur notre sol en toute impunité ? La marque Shein enregistre un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. d'euros. Pourtant, elle ne rémunère ses employés ouïghours qu'une poignée de centimes, cela bien entendu sans contrat de travail et dans des conditions on ne peut plus exécrables. Le 9 juin 2022, la veille de la Journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, le Parlement européen a cherché à protéger le peuple ouïghour en interdisant l'import de produits issus de leur travail forcé, mais sans s'en donner véritablement les Si la réalité des persécutions que subit ce peuple ne fait plus débat, si la nature même d'un génocide se profile, l'effectivité limitée des mesures européennes nous invite à vouloir aller plus loin pour pour défendre le respect des droits de l'homme. Trop d'enseignes de géants de la mode que nous avons tous fréquentées au moins une fois font des profits colossaux en vendant ces articles produits en Chine au mépris des droits de l'homme. d'avril dernier, le combat des ONG contre ces pratiques a été classé sans suite. Le besoin de nouveaux instruments apparaît évident. La proposition de résolution dont nous débattons aujourd'hui vise à assurer une meilleure traçabilité, afin qu'il soit démontré que ces produits importés ne sont pas issus du travail forcé ouïghour et que l'industrie textile, pour ne citer qu'elle, ne puisse plus se cacher derrière son ignorance. Mes chers collègues, puisque tout reste à faire, puisque des textes ambitieux sont nécessaires, apportons notre soutien à cette cause juste. Pour que l'histoire ne puisse plus tard, nous juger pour notre inaction, adoptons aujourd'hui cette résolution. Ne disons pas, plus tard, que nous ne savions pas. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires de leur initiative, qui permet la tenue de ce débat sur le triste sort de la population ouïghoure. Au lendemain des crimes contre l'humanité commis dans des camps de concentration par les régimes totalitaires d'Hitler ou de Staline, on croyait avoir tourné la page d'une telle barbarie. Eh bien non : au XXI siècle, nous devons encore déplorer des tragédies humanitaires ! Depuis maintenant plusieurs années, la République populaire de Chine bafoue les droits humains de la population ouïghoure et d'autres peuples turciques, et ce dans une certaine indifférence de la communauté internationale. Les auteurs de la proposition de résolution l'ont rappelé, les Ouïghours représentent la population chinoise musulmane, originaire du Xinjiang, une vaste région historiquement connue comme point de contact entre la Chine et le Moyen-Orient. Les faits sont très documentés : les Ouïghours sont soumis à des arrestations arbitraires, à la déportation, au travail forcé et à des violences morales et physiques. Dans les centres d'internement et d'endoctrinement où ils sont enfermés, ils subissent les pires supplices, parmi lesquels, de façon systématique, des flagellations, des électrifications, des stérilisations et avortements forcés, des viols. Comme si cela ne suffisait pas, pour que soit bien marquée la raison de cet acharnement, les Ouïghours se voient infliger des pratiques allant à l'encontre du libre exercice de leur culte, comme l'ingestion forcée de porc ou d'alcool et l'interdiction de prier. Les autorités chinoises font preuve d'une imagination terrifiante et sans borne. J'ajoute que ces atrocités n'ont pas de limite d'âge ou de genre. On dénombre, dans ces camps, environ 1 million à 2 millions de femmes, d'hommes, mais également des enfants. Séparés de leurs familles, ceux-ci sont soumis aux mêmes conditions de vie que leurs aînés, notamment en matière de travail forcé. Si ces crimes se déroulent très loin de nous, gardons à l'esprit que chaque Ouïghour de la diaspora vivant en France compte au moins un proche dans les camps de concentration, les prisons ou les usines de travail forcé du régime chinois. Selon un groupe d'avocats et d'experts des droits humains, il s'agit d'un véritable génocide, car les autorités chinoises, comme on le sait, souhaitent éradiquer une population en raison de sa confession et la rééduquer aussi bien culturellement que politiquement. Face à cela, que pouvons-nous faire ? Sans aucun doute, dénoncer et boycotter les multinationales, comme le groupe français SMCP, qui détient Sandro,

Leurs succès commerciaux ont le goût du sang, tant ils nient les principes de l'OIT, qui condamnent l'esclavage, le travail forcé, le travail des enfants, toutes formes de discrimination raciale, de torture et de châtiments cruels. Faut-il rappeler aussi l'article 33 de la Constitution de la République populaire de Chine, qui énonce que l'État « respecte et garantit les droits de l'homme Au mépris de son propre texte fondamental et des textes fondateurs du droit humanitaire international, l'État chinois commet en toute impunité ces crimes, avec la complicité des grandes multinationales. La communauté internationale, dont la France, dont la France, toujours écoutée en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a le devoir de protéger la population ouïghoure. Cela fera bientôt deux ans que les États-Unis ont promulgué un texte de loi loi interdisant l'achat de produits qui seraient fabriqués en partie ou totalement dans le Xinjiang. De son côté, l'Europe avance timidement, ménageant la Chine- disons-le -pour les raisons économiques et diplomatiques que nous connaissons. Toutefois, regardons comment la Russie nous rend la bienveillance que nous avions toujours eue à son égard jusqu'à la veille de son agression contre l'Ukraine ... La peur de contrarier n'évite pas le danger Dans ces conditions, la France doit s'impliquer pour la mise en place d'un embargo européen strict sur les produits issus du travail forcé. Le dispositif de la Commission européenne doit être revu en faveur d'un dispositif clair et opérationnel, bloquant aux frontières les importations entachées de sang ouïghour. Ainsi, le groupe RDSE approuve la proposition de résolution et la votera. La parole

monsieur le ministre, mes chers collègues, en dépit de ses dénégations obstinées, malgré la chape de plomb qu'il fait peser sur tout un pays, et spécialement sur ses provinces situées à l'ouest, le régime chinois ne parvient plus à dissimuler la nature de ses agissements contre la minorité ouïghoure. Depuis plusieurs années, en effet, les témoignages de persécutions qui nous parviennent de la région du Xinjiang sont à la fois de plus en plus nombreux, de plus en plus précis, mais aussi de mieux en mieux étayés par une pluralité d'enquêtes et de rapports internationaux. Surveillance généralisée, restrictions religieuses et linguistiques, arrestations arbitraires, internements de masse, travail forcé, viols systématisés, stérilisations, torture : la gravité des accusations qui pèsent sur Pékin est accablante. À ce jour, leur qualification exacte fait encore l'objet de nombreux débats d'experts. Mais, qu'on la nomme « violations graves des droits fondamentaux », « crimes contre l'humanité » ou bien « génocide », la réalité du supplice vécu par les Ouïghours, elle, ne peut plus raisonnablement être mise en doute. Face à ce constat, qui s'impose chaque jour avec davantage de force, la réaction internationale se distingue pourtant par sa retenue. Le récent rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a matérialisé une prise de conscience réelle sur le sujet. Mais la polarisation du monde, conjuguée à la prépondérance croissante de la Chine dans toutes les dimensions des relations internationales, risque d'entraver encore longtemps la réponse des instances multilatérales. D'autres moyens d'action doivent donc être explorés. L'Union européenne a ainsi décidé, en 2021, conjointement avec d'autres pays occidentaux, de hausser le ton et d'adopter des mesures restrictives. Ces sanctions, les premières visant la Chine depuis Tiananmen, ont constitué un signal politique et diplomatique majeur, qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais, en se contentant de geler les avoirs d'une poignée de responsables chinois et de leur interdire de pénétrer sur le territoire européen, leur ampleur apparaît, il est vrai, bien modeste au regard des faits incriminés. Il était donc important que la réponse européenne puisse franchir une nouvelle étape, mais aussi qu'elle dépasse le seul terrain diplomatique, pour viser également le champ des échanges commerciaux, fondement de la puissance chinoise. Nous savons tous combien notre relation à la Chine, et tout particulièrement notre relation commerciale, est un sujet délicat, sur lequel les sensibilités et les intérêts des États membres ne s'alignent pas spontanément. Très attendue, la proposition de règlement européen sur l'interdiction des produits issus du travail forcé est donc, à ce titre, une initiative qui mérite d'être saluée et soutenue. Certes, le projet de texte ne vise pas spécifiquement la Chine, puisqu'il prévoit que tous les biens issus du travail forcé devront être bannis du marché européen, et ce quelle que soit leur provenance. du travail nous rappelait encore récemment que près de 28 millions de personnes, sur les cinq continents, étaient touchées par cette forme d'esclavage moderne. Néanmoins, ce large cadre géographique ne devrait pas empêcher l'Europe de cibler ses efforts contre le travail forcé. En effet, les autorités chargées d'appliquer la législation devront adopter une approche fondée sur les risques. En d'autres termes, elles devront orienter leurs investigations en priorité vers les zones et les secteurs présentant les plus forts risques de travail forcé. Pour ce faire, elles devront prendre en compte les informations émanant de nombreuses sources, telles que les témoignages individuels, les éléments communiqués par les ONG ou encore les données recueillies auprès des entreprises, notamment dans le cadre de l'exercice de leur devoir de vigilance. Les autorités pourront en outre s'appuyer sur les travaux de leurs homologues européens, réunis au sein d'un nouveau réseau contre les produits issus du travail forcé, ainsi que sur les orientations fournies par la Commission européenne au travers des lignes directrices, des indicateurs de risques et de la base de données qu'elle publiera. Ainsi, dans la pratique, et au vu de la somme d'informations déjà collectées à ce jour, l'application de ce dispositif aboutira inévitablement à placer le Xinjiang et ses exportations au sommet de la liste des enquêtes à mener par les autorités nationales. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui suggère néanmoins une approche différente de celle que préconise la Commission. Dans un premier temps, ses auteurs invitent l'Union européenne à renforcer ses sanctions contre les auteurs des crimes perpétrés contre contre la communauté ouïghoure. Je crois que nous pouvons tous, sur ce point, nous retrouver et considérer que les mesures actuellement en place méritent d'être à la fois approfondies et élargies. Dans un second temps, il est proposé d'introduire, au sein du projet de règlement européen, un régime spécifique à la région du Xinjiang. Selon les termes de l'exposé des motifs, il s'agirait de mettre en place un embargo sur les produits issus du travail forcé de la population ouïghoure. Comment, là encore, ne pas souscrire à un tel objectif ? Le système proposé par nos collègues me laisse, en revanche, plus dubitative. En effet, celui-ci s'inspirerait du mécanisme qui est mis en oeuvre depuis un an par les États-Unis et qui prévoit que les marchandises en provenance du Xinjiang sont automatiquement réputées enfreindre l'interdiction de travail forcé, sauf à ce que l'importateur puisse prouver le contraire d'une manière « claire et convaincante Dès lors, avec le texte qui nous est proposé, il appartiendrait non plus aux autorités de prouver une infraction, mais aux entreprises de démontrer son absence, qui plus est « hors de tout doute Disons-le d'emblée : dans le labyrinthe des chaînes d'approvisionnement modernes, éliminer ce doute sera quasiment impossible, tant il est complexe pour une entreprise, et spécialement pour une PME, de connaître l'ensemble des acteurs participant à la fabrication d'un produit. À ce titre, il est important de souligner que si l'enchevêtrement des chaînes de valeur peut se révéler un obstacle infranchissable pour les entreprises, la proposition de règlement européen fait en sorte qu'il n'en soit pas de même pour les autorités. En effet, celles-ci pourront interdire la commercialisation d'un produit même si tous les éléments prouvant qu'il est issu du travail forcé n'ont pas pu être réunis. Dans ce contexte, une inversion de la charge de la preuve n'apparaît pas véritablement indispensable. Surtout, en raison de la responsabilité exorbitante et des risques de non-conformité qu'elle ferait peser sur les entreprises, une telle mesure risque de les inciter à se désengager de toute activité en lien avec le Xinjiang. L'exemple américain nous fournit d'ailleurs un précédent instructif, puisque nombre d'entreprises, américaines ou non, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles cesseraient purement et simplement de s'y approvisionner, afin de maintenir leur accès au marché américain et d'éviter tout risque de sanction. À À la lumière de cet exemple, il est à craindre que l'embargo proposé par nos collègues sur les produits du travail forcé des Ouïghours ne se transforme en embargo tout court, privant ainsi toute la province d'une grande partie des débouchés sur lesquels repose actuellement son activité économique. Je crois donc qu'il faut aussi et peut-être avant tout mesurer pleinement les effets secondaires que pourrait avoir un tel embargo sur la population du Xinjiang, donc sur les Ouïghours eux-mêmes. Plus largement, chacun a pris conscience ces dernières années que la traçabilité et la responsabilisation des chaînes d'approvisionnement étaient désormais des impératifs incontournables. Mais il m'apparaît essentiel sur ce sujet d'éviter les ruptures et d'avancer pas à pas. essentiel d'adopter une logique partenariale entre des États légitimement de plus en plus exigeants et des entreprises de plus en plus mises à contribution, mais aussi- il faut le souligner -de plus en plus engagées. C'est pourquoi, même si nous comprenons l'objectif de ce texte, le dispositif proposé ne nous semble pas le plus opportun. Le groupe Les Républicains s'abstiendra donc sur cette proposition de résolution. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec son développement économique spectaculaire et ses prouesses technologiques, nous pourrions presque oublier que la Chine est communiste. L'enfer des camps nous le rappelle. Depuis la fin du XX siècle, et plus encore depuis 2014, le parti communiste chinois emploie les grands moyens pour régler son problème ouïghour. Cette minorité ethnique de 11 millions de personnes est la cible d'une persécution génocidaire. Sous couvert de lutte contre l'islamisme, les dirigeants chinois enferment à grande échelle cette population. Dans la droite ligne totalitaire communiste, le parti organise la rééducation des individus à travers un système concentrationnaire. Avec sa discipline de fer, il tente de briser les consciences et la croyance religieuse par l'endoctrinement. Le marxisme n'ayant jamais été très convaincant, le parti recourt volontiers aux séances de torture, aux viols et au travail forcé. La rééducation, criminelle en elle-même, n'est cependant qu'une façade. Pour régler le problème, les autorités chinoises entreprennent de le faire disparaître. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU les accuse ainsi de procéder à des campagnes de stérilisation forcée. L'objectif est d'effacer la culture ouïghoure, la langue ouïghoure, mais aussi la minorité ouïghoure dans son ensemble. Ces actes portent atteinte à l'humanité et déshonorent la Chine millénaire. Ils appellent la plus ferme condamnation. C'est le sens du présent texte déposé par le groupe Écologiste -Solidarité et Territoires. Sans se contenter de saluer l'initiative de nos collègues, notre groupe a cosigné cette résolution à l'unanimité. Le martyre des Ouïghours n'est- hélas ! -pas un cas isolé. Avant eux, il y a déjà eu tous ceux qui furent décrétés nationalistes, contre-révolutionnaires, comme les militants des droits humains ou encore les Tibétains. 50 millions de personnes qui sont passées par les camps du parti ; 20 millions de personnes y sont mortes. Ce n'est pas un hasard si la Chine a toujours eu recours à l'emprisonnement de masse. Comment pourrait-il en être autrement quand hors de la majorité ne peuvent se trouver que les ennemis du peuple ? La réalisation du bien commun implique la surveillance et le contrôle des individus. Il faut s'assurer de leur obéissance et les priver des moyens de s'opposer. Ainsi disparaissent le droit de propriété et la liberté. Un tel système carcéral coûte cher. Pour le maintenir, les autorités chinoises équilibrent les finances en recourant au travail forcé. Aujourd'hui comme hier, les détenus travaillent sans relâche entre les séances de torture et d'autocritique. Les marchandises issues du travail forcé sont souillées du sang des victimes du régime communiste. Défenseurs de la liberté, nous ne pouvons pas commercer avec ses fossoyeurs. La résolution propose que ces biens ne franchissent pas nos frontières ; nous ne pouvons que l'approuver. Par sa cosignature et par son vote à l'unanimité, le groupe Les Indépendants affirme son opposition à toutes les oppressions. Les Ouïghours, comme toutes les minorités, comme tous les individus, ont droit au respect de leur liberté. La parole

délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je mesure la gravité du sujet qui m'amène aujourd'hui à prendre la parole devant vous à l'occasion de l'examen de cette proposition de résolution visant à interdire l'importation des produits issus du travail forcé de la population ouïghoure en République populaire de Chine. Depuis plusieurs années, la situation des droits de l'homme au Xinjiang fait l'objet des plus vives préoccupations. Des témoignages et des rapports étayés ont notamment fait état d'internements de masse et de détentions arbitraires, de disparitions forcées, de violences sexuelles, de surveillance généralisée ainsi que de travail forcé, sujet au coeur de la proposition de résolution examinée aujourd'hui. Ces informations ont été confirmées par les conclusions du rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Xinjiang, publié en août 2022. Celui-ci souligne également que l'ampleur de la détention arbitraire et discriminatoire subie par les personnes ouïghoures et d'autres groupes à prédominance musulmane pourrait être constitutive de crimes internationaux, en particulier de crimes contre l'humanité.

estimait en juillet 2022 pouvoir raisonnablement conclure que des Ouïghours, des Kazakhs et des membres d'autres minorités ethniques avaient été soumis au travail forcé dans des secteurs tels que l'agriculture et l'industrie manufacturière dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, en Chine. Face à la gravité de la situation au Xinjiang, la France est pleinement mobilisée à tous les niveaux. Tout d'abord, dans le cadre du dialogue étroit et exigeant qu'elle mène avec la Chine, la France évoque les droits de l'homme en Chine, en particulier au Xinjiang, lors des entretiens bilatéraux jusqu'au plus haut niveau. Nous relayons auprès des autorités chinoises nos préoccupations, partagées par l'opinion publique française, quant à l'ampleur et à la gravité des violations au Xinjiang, et appelons à y mettre fin. Le Président de la République s'est lui-même à plusieurs reprises exprimé publiquement avec force à ce sujet. L'ambassade de France en Chine poursuit, en dépit d'un contexte difficile, son action de soutien à la société civile et aux militants des droits de l'homme. S'agissant de notre territoire national, les autorités françaises sont très attentives au respect des droits fondamentaux des Ouïghours établis en France, ainsi qu'à leur sécurité, comme elles le sont pour toutes les personnes présentes sur notre territoire, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère. Au niveau européen, notre action a pris une dimension nouvelle avec l'adoption de sanctions, le 22 mars 2021, au titre du régime transversal de sanctions de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Parmi les personnes et entités sanctionnées, quatre individus et une entité ont été désignés pour leur responsabilité dans les violations des droits de l'homme perpétrées au Xinjiang. Ces mesures constituaient une première depuis les sanctions adoptées en 1989. Le Xinjiang a également été l'objet d'échanges approfondis à l'occasion de la 38 session du dialogue Chine-Union européenne sur les droits de l'homme

Cette vigilance européenne a eu des résultats, avec la ratification par la Chine des conventions fondamentales n 29 et 105 de l'OIT sur le travail forcé. Bien entendu, au-delà de la ratification, la question de la mise en oeuvre de ces conventions est toujours présente dans nos échanges avec Pékin. Par ailleurs, comme vous le savez, le processus de ratification de l'accord sur les investissements est interrompu depuis que la Chine a sanctionné des élus et des parlementaires, en particulier des parlementaires européens. ce qui concerne les enceintes internationales, la France y soutient systématiquement les déclarations et les résolutions dénonçant la situation au Xinjiang, prononcées au sein de la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil des droits de l'homme Ainsi, le 6 octobre dernier, lors de la 51 session du CDH, la France a appelé à tenir un débat à la suite de la publication du rapport du HCDH sur la situation des droits de l'homme dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Après vous avoir exposé les différents piliers de notre politique en matière de droits de l'homme au Xinjiang, je voudrais en revenir au sujet de la lutte contre le travail forcé et au devoir de vigilance des entreprises. L'engagement de la France dans ce domaine est, vous le savez, pionnier. est en effet le premier au monde à s'être doté, dès 2017, d'une loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Cette loi vise à identifier les risques liés aux activités des entreprises et à leurs chaînes de valeur afin de prévenir et d'atténuer les atteintes graves aux droits fondamentaux, y compris le travail forcé et les atteintes Elle impose aux entreprises d'établir un plan de vigilance, inclus dans le rapport de gestion de l'entreprise. Nous conduisons à cette fin des actions de sensibilisation, afin de veiller à ce que le secteur privé prenne sa part de responsabilité pour lutter contre le travail forcé. Notre objectif aujourd'hui est que l'Union européenne prenne des mesures à la hauteur des enjeux. C'est pourquoi la France a fait du capitalisme responsable une des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022. Dans ce cadre, elle a pris une part active à l'élaboration du projet de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, présenté par la Commission en février 2022. La France continue de mettre son expérience, accumulée grâce à sa loi nationale, au service de la négociation en cours. Elle participe également activement aux travaux menés en vue d'adopter un règlement pour interdire à tous les opérateurs économiques la mise sur le marché européen de produits issus du travail forcé, qu'ils soient fabriqués sur le territoire de l'Union européenne ou importés, ainsi que l'exportation de tels produits depuis l'Union européenne. La France sera donc attentive à ce que le projet de règlement soit davantage clarifié pour garantir son opérationnalité et sa prévisibilité, tant pour les entreprises que pour les autorités chargées de son application. Nous appelons à ce que les discussions européennes s'accélèrent aujourd'hui sur le sujet. En outre, notre pays déploie son action à l'échelle mondiale et multilatérale pour lutter contre le travail forcé. Il promeut le développement, la ratification et l'application effective des normes internationales pour interdire le travail forcé. L'entrée en vigueur pour la Chine des conventions fondamentales n 29 et 105 de l'OIT sur le travail forcé, cet été, déclenchera les mécanismes de suivi et de contrôle qui sont prévus pour ces conventions. La vigilance du Gouvernement s'exerce aussi en matière de financement du développement. Nous contestons tout financement, y compris par l'intermédiaire des banques de développement, de projets susceptibles de contribuer au travail forcé ou à la répression, notamment dans la région du Xinjiang. La France tient aussi un rôle moteur au sein de l'Alliance 8.7, partenariat mondial pour l'éradication du travail forcé, de l'esclavage moderne, de la traite des êtres humains et du travail des enfants dans le monde. Dans le cadre du G7, la France a signé plusieurs déclarations politiques visant à réaffirmer son engagement à lutter contre le travail forcé à l'échelle mondiale, la plus récente étant celle signée à Hiroshima le 20 mai 2023. La France est aussi très active dans la négociation et les discussions relatives à la conduite responsable des entreprises au sein de l'OCDE, qui est l'enceinte de référence en la matière, ayant permis d'élaborer des bonnes pratiques et des outils concrets à l'intention des entreprises. Ces différents exemples témoignent de l'engagement de la France sur la thématique du travail forcé au niveau tant national, européen qu'international. Vous aurez constaté une grande convergence entre l'action du Gouvernement et les recommandations contenues dans cette proposition de résolution parlementaire. Le travail forcé constitue toutefois un problème d'ampleur mondiale que l'on ne saurait circonscrire à une seule région. C'est pourquoi nous défendons le principe d'une réponse mondiale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la France continuera de mener avec ses partenaires européens un dialogue exigeant et- disons-le -difficile avec la Chine sur le respect des droits de l'homme, notamment au Xinjiang, en appelant en particulier la Chine à ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies. Nous poursuivrons par ailleurs, sans relâche, notre engagement afin que soient bien pris en compte les objectifs fixés au niveau européen en matière de respect des droits de l'homme en Chine, en particulier au Xinjiang et dans le cadre de la politique commerciale et d'investissement. Dans les instances internationales, nous demeurerons pleinement mobilisés afin de défendre le caractère universel et inaliénable des droits de l'homme et d'exhorter la Chine à respecter ces libertés fondamentales, conformément à ses obligations découlant du droit national et international. La discussion